sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19, en application de l'article 50-1 de la Constitution.

La situation sanitaire reste préoccupante, et nous avons atteint depuis une dizaine de jours un plateau, qui se situe malheureusement à un niveau ne permettant pas encore de garantir une pleine maîtrise de la circulation virale, alors même que les fêtes de fin d'année approchent. La deuxième vague n'est pas derrière nous. Aussi, la prudence et la vigilance devront rester de mise pendant de longues semaines encore. L'arrivée du vaccin et le lancement dans notre pays de la campagne vaccinale dans les toutes prochaines semaines constituent cependant un grand motif d'espoir. Le Gouvernement a souhaité préciser au Parlement les fondements de notre stratégie vaccinale et ses modalités de mise en oeuvre, mais aussi la façon dont il l'intègre à son dispositif global de lutte contre le virus. Il est essentiel que nous puissions, ensemble, engager un débat constructif sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle, au-delà de cette séance, un cadre de dialogue pérenne a été installé, avec la mise en place d'un comité permanent comprenant les présidents de chacune des assemblées et les présidents de l'ensemble des groupes parlementaires.

Je sais que nous serons collectivement à la hauteur. Depuis le début de cette crise sanitaire, le Sénat a été une force motrice. Les territoires, les collectivités territoriales, les élus locaux ont, eux aussi, été en première ligne face à la détresse de nos concitoyens. Dès le printemps dernier, la France a pris l'initiative de demander la création d'une européenne capable de constituer une seule force d'achat, de façon à peser dans les négociations et à éviter une compétition nécessairement contre-productive entre les pays européens.

À ce stade, les vaccins les plus avancés sont ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna. D'autres vaccins se situent en phase 3 des essais cliniques et pourraient être disponibles dans les mois qui viennent.

Des précisions seront fournies dans un avis complémentaire de la HAS sur les autres structures qui accueillent des personnes âgées et qui, sans être spécialisées dans l'accueil de ces dernières, pourraient également être concernées par cette première étape.

Cette première étape sera décisive, mais les personnels des établissements pour personnes âgées ne seront pas seuls pour la franchir- je m'y engage. Ils seront informés à l'avance et les Agences régionales de santé, les ARS, se tiendront à leurs côtés pour que l'approvisionnement se déroule dans les meilleures conditions.

nous demanderons aux équipes soignantes de ces établissements de rechercher le consentement de la famille. Cela prendra forcément un peu de temps, chacun peut le comprendre.

les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique- la sécurité, l'éducation ou encore l'alimentation -, les personnes vulnérables et précaires, ainsi que les professionnels qui les prennent en charge, les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos, puis le reste de la population majeure. Pourquoi

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes bel et bien entrés dans l'organisation de la campagne vaccinale. C'est une véritable épreuve logistique, tant l'échelle est sans comparaison avec nos habitudes en la

Pour relever ce défi, nous avons fait le choix de la compétence et de la connaissance, en nous appuyant sur les pharmaciens et les circuits logistiques de transport de médicaments sensibles et en renforçant encore la sécurisation de toutes les étapes, partout où cela faisait sens.

est issu d'une start-up allemande, qui a conclu un partenariat avec un groupe pharmaceutique américain pour pouvoir produire plus massivement dans le monde. Le site de production des vaccins qui seront distribués aux Français est situé en Belgique, donc pas très loin de chez nous.

je ne crois pas que nous pourrons créer l'adhésion des Français sur la vaccination- vous savez combien nos concitoyens sont exigeants sur ce sujet -sans nous appuyer sur les communautés médicales, paramédicales et scientifiques. Toutefois, je sais aussi que nous serions peu de chose

la confiance est un élément très important ! Le Gouvernement a aussi saisi le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, pour mettre en place un collectif de citoyens chargé d'émettre des observations et de formuler des recommandations sur la politique conduite.

matière -ou pour mettre en place ce programme opérationnel de vaccination. Je dois le dire, l'Europe s'est montrée unie, soudée et ambitieuse pour préparer de manière efficace et à grande échelle cette campagne vaccinale historique. Avec mes homologues allemand, belge, espagnol, italien, luxembourgeois, néerlandais, mais également suisse,

L'annonce d'une campagne de vaccination par la présidente de la Commission européenne le 16 décembre dernier, campagne qui commencera le même jour dans tous les pays de l'Union européenne, est une immense source d'espoir.

vaccinées seront ou non passibles de transmettre le virus sous une forme bénigne ou grave, ce qui, jusqu'à présent et avec d'autres vaccins, n'existait jamais, sauf, me semble-t-il, pour le vaccin contre la poliomyélite. Il nous faudra marteler que ces campagnes de vaccination, longues et ciblées, seront couronnées de succès si, dans le même temps, nous continuons à pratiquer le port efficace du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Cependant, dans le contexte bien français de défiance à l'égard des vaccins, alors que le vaccin ARN messager n'a pas d'adjuvant,

de deux doses -, l'action de ciblage des populations encouragée par la Haute Autorité de santé est nécessaire, mais elle méritera elle aussi une communication convaincante et répétée. Le choix des Ehpad, guidé par un objectif de protection d'une population hyperfragile, semble judicieux, mais comment communiquer sur le fait que les résidents des Ehpad y restent statistiquement au maximum entre deux ans et demi et trois ans ? ? Comment expliquer que les personnes mourant dans ces établissements dans les jours ou mois suivant la vaccination ne décéderont pas de cette Il a été décidé aussi que les personnels soignants présentant des maladies graves et ceux qui sont volontaires seront vaccinés prioritairement. C'est évidemment indiscutable, et il semble que ces patients soient, pour la plupart d'entre eux, demandeurs de cette vaccination. Toutefois, des personnes âgées valides demeurant chez elles, qui ont déjà subi deux confinements, et qu'il faudrait vacciner rapidement pour leur permettre de reprendre une vie sociale, source d'équilibre physique et psychique ? . Eh oui ! Sinon, rapidement, nous aurons affaire à une nouvelle vague de décès de personnes âgées, cette fois due à l'isolement et au syndrome de glissement. Ce qui a été dit lors des auditions qui ont été réalisées par la commission des affaires sociales, c'est que ce vaccin protégerait contre les formes malignes et bénignes de la maladie, mais qu'il existe une incertitude sur la transmission, d'où la non-vaccination des jeunes en priorité. Il est donc important, en attendant des études plus poussées sur ces vaccins ARN et les autres vaccins plus conventionnels- leurs retards sont probablement un peu le reflet de la façon dont, en France, on traite les innovations

J'aimerais en venir maintenant à un point qui me tient à coeur, monsieur le ministre. Si j'ai bien compris, les laboratoires français ont négligé la recherche sur les vaccins à ARN messager, ARN messager, biotechnologie pourtant utilisée dans d'autres domaines de la santé, en particulier en cancérologie, avec succès et sans intolérance pour les patients soignés de cette façon. Si je cherche à savoir pourquoi, je n'ai pas de réponse idéale, sauf que, me semble-t-il, la France, comme on le voit sur d'autres types de recherche, en particulier en bioéthique, est frileuse dès qu'il s'agit de financer des travaux, qui, pour la plupart d'entre eux, n'aboutiront pas. pas. Les chercheurs ou les projets partent donc vers des cieux plus cléments, avec des chances de succès beaucoup plus grandes ... Il est tout de même dommage de constater que notre pays est absent sur la technologie de l'ARN messager. Il faudra, la lumière de cette aventure supplémentaire, revoir notre système de pensée sur le financement de la recherche. Pour ma part, je n'aurais pas honte de mettre en place des cofinancements public et privé.

Le Premier ministre a déclaré jeudi dernier que « c'est en France que la situation est aujourd'hui la mieux maîtrisée par rapport à nos voisins ». La semaine dernière, le taux d'incidence de la covid y était de 107 pour 100 000, contre 143 en Belgique, 150 en Allemagne et 250 en Suisse. 10 000 cas quotidiens en France, contre 30 000 en Allemagne. Il faut se pincer pour y croire ! Cependant, ces chiffres sont précaires, et après avoir fait pendant huit mois un complexe d'infériorité vis-à-vis des Allemands, ne faisons surtout pas aujourd'hui un complexe de supériorité. Ce virus continue d'être méconnu, déroutant et traître. Sauf, bien sûr, pour ceux qui ont une boule de cristal. Lors du déconfinement, en mai dernier, j'avais taclé le professeur Mélenchon, de la faculté de médecine de La Havane, qui avait annoncé, à l'Assemblée nationale, l'arrivée inéluctable d'un deuxième pic de l'épidémie. Au même moment, son collègue, le professeur Raoult, de la faculté de médecine de Marseille, annonçait avec la même certitude qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Bingo ! C'est Mélenchon qui a décroché le pompon et qui s'est immédiatement auto-décerné sur Twitter le prix Nobel de médecine prophétique, comme tant d'autres, d'ailleurs, sur les plateaux de télévision. Je n'ai rien à changer à ce que j'ai dit à l'époque : on a parfois une chance de tomber juste en jouant à Paul le poulpe. Après tout, même les horloges arrêtées donnent l'heure exacte deux fois par jour. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les complotistes ont tort. Tous les anti-science sont en train de recevoir le meilleur des démentis, et les scientifiques la meilleure des confirmations : 7 jours en janvier dernier pour séquencer le génome du virus 303 jours entre le premier patient et la sortie d'un vaccin, là où il fallait dix ans auparavant. D'ici à quelques mois, la pandémie sera vaincue par une extraordinaire performance scientifique, technologique, industrielle et logistique mondiale- j'allais dire mondialisée, mais je ne voudrais choquer personne Bien sûr les anti-science ne vont pas lâcher le morceau. Ils essaient maintenant de discréditer les vaccins, avec un certain succès si l'on en croit les sondages, qui affirment que 60 % de la population serait réticente. Les sondages disaient aussi qu'Hillary Clinton serait élue contre Trump et que les Anglais voteraient contre le Brexit Si l'on faisait le travail correctement, en demandant à ceux qui hésitent s'ils font parce qu'ils sont contre les vaccins ou parce qu'il y a encore des incertitudes, on découvrirait que les Français, loin d'être des obscurantistes, sont, au contraire, des gens très rationnels. une petite minorité d'anti-vaccins et une grande majorité qui se dit : « Avant que ma grand-mère ne se fasse vacciner, je veux être sûr qu'elle ne risque rien. » Je vais vous proposer le sondage de l'Institut Malhuret. Depuis plus d'un mois, nous sommes en rupture de stock de vaccins antigrippe. Pourtant, les laboratoires en ont produit une fois et demie plus que l'an dernier. Les pharmacies ont été dévalisées. Tout à fait ! Conclusion : quand on propose aux Français un vaccin connu et sûr, ils se précipitent dessus, surtout quand on risque, le même hiver, d'attraper la grippe et la covid. le suivant : quand nous commencerons la vaccination, après que les Anglais et les Américains l'auront expérimentée depuis un mois, ce qu'il faut craindre, c'est non pas que les doses restent dans les congélateurs, mais que nous peinions à répondre à la demande. Il y a beaucoup d'autres bonnes nouvelles en ces temps de morosité où, en plus, les jours raccourcissent : les progrès impressionnants des équipes médicales, qui ont divisé par deux les décès en réanimation le financement européen commun d'un plan de relance de 750 milliards d'euros ; la résistance de nos sociétés, notamment de la nôtre, qui a été confrontée à une triple crise, sanitaire, économique et terroriste, mais qui ne craque pas. Toutefois, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'en viens aux nouvelles plus préoccupantes, la première étant que nous sommes loin d'en avoir fini avec l'épidémie. Lors du premier discours du Premier ministre, ici, en juin, je lui avais dit qu'il s'était vu confier « un à 10 000 aspirines ». C'était peut-être en dessous de la réalité. La course de vitesse a commencé, entre la probabilité d'une troisième vague, qu'il faudra réussir à maîtriser, et l'arrivée de l'immunité collective, avec l'aide du vaccin, qu'il faudra réussir à assurer. Les mois qui viennent seront le véritable de l'épidémie pour le Gouvernement, qui sera jugé sur son issue, et pour tous les Français, qui sauront à la fin s'ils font encore partie des nations qui résistent et réussissent ou des nations déclassées et reléguées en deuxième division. Le premier acte de la pandémie fut, mondialement, une immense surprise, une immense incompréhension et une immense pagaille, sauf pour les pays asiatiques déjà confrontés au problème dans le passé. Cet acte s'est terminé par la solution la plus drastique, mais la plus coûteuse à tous points de vue, à savoir le confinement strict. Le deuxième acte a commencé par le déconfinement de l'été. Nous avions fait beaucoup de progrès- nous avions les gestes barrières, les masques, les tests et la stratégie « tester, tracer, isoler mais nous n'avons pas réussi à la contenir sur le terrain. La conséquence en fut le deuxième confinement. Le troisième acte commence aujourd'hui. Si nous voulons le réussir, il faut identifier nos points faibles, et j'en vois deux principaux. L'isolement, tout d'abord, qui divise la France en deux camps : obligatoire ou non. Posée en ces termes, la question n'a pas de solution. Entre l'isolement laissé au gré de chacun, qui aboutira au même résultat qu'en octobre dernier, et l'isolement obligatoire, qui conduira nombre de nos concitoyens à refuser les tests, la solution est un isolement réellement accompagné, avec des équipes allant à domicile et de réelles possibilités d'accueil pour ceux qui ne peuvent rester chez eux. Votre déclaration et l'annonce de moyens humains accrus montrent que vous l'avez compris. C'est sur l'action que portent mes craintes. La coordination nécessaire entre tant d'acteurs, à savoir hôpitaux publics, privés, soignants libéraux, laboratoires et collectivités territoriales, n'a jamais pu être réellement assurée jusqu'à ce jour par une administration de la santé effondrée sous son propre poids et multipliant les injonctions contradictoires. Un mauvais général vaut mieux que deux bons ! » disait Napoléon. Il y a beaucoup de choses que les Français croient que le monde nous envie, mais que le monde ne nous envie pas du tout. Vous avez là un énorme défi à relever. Le second défi est la logistique, pour acheminer les vaccins jusqu'à leurs destinataires. Je disais tout à l'heure que nous sommes en rupture de stock de vaccins antigrippe. Si l'État ne peut éviter qu'un vaccin bien connu, annuel, facile à conserver, soit absent des pharmacies depuis un mois, vous comprendrez mes inquiétudes sur sa capacité à assurer la logistique d'un vaccin produit à flux tendu, conservé à-80 degrés Celsius et commandé au même moment par le monde entier. Ma crainte n'est pas que les Français ne veuillent pas se faire vacciner ; elle est qu'ils ne puissent pas le faire. Voilà votre second défi, monsieur le ministre, et je vous souhaite de tout coeur d'arriver à le relever, et il va vous falloir encore bien des boîtes d'aspirine. Cette année se termine sur une note amère, entre le deuil de ceux qui nous ont quittés, le désespoir de ceux qui ont perdu leur travail ou qui vont le perdre, l'angoisse des acteurs du monde de la culture, de la restauration, du tourisme et de bien d'autres qui n'ont qu'une envie, reprendre leur activité, mais qui ne peuvent le faire. La France déprime, et c'est bien compréhensible, mais nous serions mal avisés d'en rester à ce constat, et surtout de le noircir encore. Le, premier magazine d'information américain, titre cette semaine : « La pire année de l'histoire ». C'est faux ! Pensons à ceux qui étaient dans les tranchées de Verdun à 18 ans, à ceux qui ont eu 20 ans en 1940. Eh oui ! Rien n'explique mieux le bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire. 2020 est une épreuve, mais ce n'est qu'une épreuve, et l'humanité en a surmonté de bien plus graves. Après 2020, année de la tristesse, viendra 2021. Et grâce aux vaccins, grâce à notre respect des règles, grâce à notre solidarité, ce sera l'année de l'espoir, l'année où nous surmonterons à notre tour l'épreuve qui nous est assignée. C'est le voeu que je forme aujourd'hui.

voilà un an que le SARS-CoV-2 est apparu en Chine. La diminution des espaces naturels et le rapprochement des habitations humaines des populations d'animaux sauvages sont vraisemblablement responsables de cette pandémie, qui a mis sens dessus sens dessus dessous les sociétés mondiales. Voilà un an que nos vies ont été profondément bouleversées par ce virus, sur lequel on a tant écrit et sur le lequel on sait encore si peu de choses. Il est encore tôt pour tirer les conséquences de cette pandémie, qui est toujours notre quotidien, mais aussi notre horizon. Cet horizon, depuis le premier confinement, seul un hypothétique vaccin semblait en mesure de nous permettre de le dépasser. Il y a un mois, alors que le Président de la République envisageait encore un vaccin à l'été, deux laboratoires annonçaient assez soudainement des résultats très encourageants, résultats très encourageants, reposant sur une méthode révolutionnaire : des vaccins génétiques s'appuyant sur l'ARN messager. Alors que la Haute Autorité de santé, la HAS, et l'Agence européenne des médicaments n'ont pas encore validé les résultats des laboratoires, des milliards de doses ont déjà été commandées par les pays européens, partout dans le monde. Vous préparez déjà la vaccination massive des Français au 1 semestre 2021. Nos voisins outre-Manche n'ont même pas attendu l'avis de l'Agence européenne et ont déjà commencé leur campagne de vaccination Il faut dire que l'impatience est grande. Le vaccin est une lumière au bout du tunnel, l'espoir du retour à la normale, de la sortie du confinement, de la réouverture de tous les lieux de convivialité, de tous les lieux culturels et sportifs, du retour au lien social. au lien social. Un troisième confinement est une perspective épouvantable d'un point de vue humain, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue économique et social, d'un point de vue financier, d'un point de vue global Monsieur le ministre, vous jonglez avec les injonctions contradictoires, cherchant le bon chemin pour sortir du maquis ; nous le savons. Il n'en demeure pas moins que tout ceci est vertigineux. On s'apprête à inoculer à des milliards d'êtres humains un vaccin révolutionnaire, produit dans un temps record, avec des essais cliniques largement raccourcis, le tout pour prévenir une maladie que nous connaissons encore mal. Même si le ratio bénéfices-risques des vaccins sur le marché justifie largement la stratégie de vaccination rapide que vous nous proposez, les raisons de l'inquiétude sont légitimes, et il ne faut surtout pas les balayer du revers de la main. Ainsi, 60 % de nos compatriotes n'envisagent pas de se faire vacciner. Au pays de Pasteur, une telle enquête fait frémir, et il faut absolument en envisager toute la portée, car aucune des stratégies de vaccination que vous pourrez imaginer ne fonctionnera sans l'assentiment des Françaises et des Français. Vous tentez de répondre aux inquiétudes en instaurant ce conseil citoyen, présidé par l'incontestable Alain Fischer. Le Sénat s'est ému, à juste Le Sénat s'est ému, à juste titre, de la multiplication des structures pour organiser les solutions face à la crise, mais, pour le coup, la défiance étant telle, à votre endroit comme au nôtre, qu'une instance citoyenne semble indispensable pour reconstruire un tant soit peu de confiance- à condition de ne pas la substituer à la représentation nationale, bien sûr. Tel ne semble pas être le cas, puisque vous sollicitez le Parlement en amont, et nous saluons cette évolution, comme nous saluons la multiplication des réunions d'information et de concertation. Il faut poursuivre dans cette voie. En matière de confiance, la transparence est le maitre mot, et je fais miennes les recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : publier sur une plateforme unique en version complète, comme en version synthétique, l'intégralité des informations disponibles sur tous les vaccins proposés prévenir tout conflit d'intérêts, en rendant obligatoire la publication de la déclaration d'intérêts de toutes celles et tous ceux qui officient à l'élaboration et au déploiement de la stratégie vaccinale. J'en ajouterai une troisième, indispensable : la publication des contrats signés par l'Union européenne avec les laboratoires pharmaceutiques. reconstruire la confiance dans un temps si court ne passera, hélas, certainement pas uniquement par les pouvoirs publics. Tout au plus, en agissant ainsi, vous pouvez éviter d'aggraver la défiance. Reconstruire la confiance passera par les liens humains, par les médecins généralistes et, demain, on l'espère, par les pharmaciens. Tant que le vaccin, celui de Pfizer pour ne pas le nommer, nécessitera une telle logistique et une telle chaîne du froid, malheureusement, il sera difficile de s'appuyer sur ces relais de proximité en lesquels nos concitoyennes et nos concitoyens ont confiance,

Globalement, la stratégie que vous nous proposez, notamment son phasage, nous apparaît bien calibrée. Nous vous invitons à ne pas précipiter les choses, si d'aventure les conclusions de l'Agence européenne et de la HAS étaient mitigées, ou si vous rencontriez des difficultés logistiques à même de perturber le lancement de la première Cette stratégie de phasage permettra de cibler les publics et de se prémunir d'une pénurie, comme nous en connaissons actuellement avec le vaccin de la grippe. Par ailleurs, sur recommandation, notamment de l'épidémiologiste Alfred Spira, nous vous demandons de bien vouloir permettre, dès la première phase, la vaccination de certains publics particulièrement fragiles et exposés les personnes vivant en foyer de travailleurs migrants. Il s'agit de personnes souvent âgées, présentant une forte fragilité sanitaire et de fréquents problèmes de vulnérabilité psychique. En situation de séjour régulier, elles connaissent pourtant d'importantes difficultés financières, vivent en collectivité et dans une grande promiscuité. également les personnes porteuses d'affections psychiatriques chroniques vivant en institution de moyen et long séjour, particulièrement fragiles et fortement touchées matériellement et socialement par la crise.

Il paraît cohérent de les vacciner, s'ils le souhaitent, dès la deuxième phase, à la même période que les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social qui les suivent. Enfin, nous saluons votre décision de prendre en charge intégralement le coût des vaccins. Nous vous demandons en complément de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes les plus précaires n'aient pas de frais à avancer. Nous n'avons encore que très peu de recul sur ces vaccins, mais ils mais ils semblent protéger efficacement les personnes les plus exposées à la violence du virus, sans présenter de risques ou d'effets secondaires handicapants. La transparence doit bien sûr toujours rester Cependant, ce vaccin n'est pas le bout du tunnel que je décrivais tout à l'heure. Nous n'avons encore aucune certitude sur le fait qu'il bloque totalement la transmission du virus. Aussi, s'il permet, nous le souhaitons, aux secteurs les plus touchés par les mesures de confinement de reprendre progressivement leur activité, il ne doit surtout pas apparaître comme un « totem d'immunité », pour reprendre vos mots, monsieur le ministre. Le chemin est encore long pour sortir de cette épreuve et, pourtant, nous avons terriblement besoin de retrouver un peu de nos vies en dehors de l'activité économique. C'est votre défi, dans la période qui s'ouvre : reconstruire cette confiance ; rééquilibrer les mesures coercitives qui perdureront contraindre davantage le travail pour permettre la reprise des autres activités humaines. Dans cette période incertaine, notre population est épuisée et a besoin de perspectives rapides, d'oxygénation mentale, que le vaccin n'apportera pas dans un futur proche. Il faut permettre de supporter l'incertitude. Comme le dit Edgar Morin, « l'incertitude contient en elle le danger, et aussi l'espoir.

Dix mois après le début de cette pandémie sans précédent, à l'heure où des campagnes de vaccination se mettent en place aux quatre coins du monde, le Gouvernement présente les principaux volets de la stratégie vaccinale française et sa place dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19. Il est heureux que nous ayons ce débat. En effet, avec un calendrier si rapide qu'il impressionne autant qu'il interroge, nous nous devons de proposer aux Français une discussion constructive sur les axes qui le guident. La méfiance et le scepticisme peuvent être compréhensibles. Aussi, il nous faut continuer à restaurer la confiance et construire l'adhésion au vaccin autour de quatre principes. Le premier principe est le libre choix : le Président de la République l'a dit, la vaccination ne sera pas obligatoire. Pour autant, nous espérons que la défiance à l'égard de celle-ci sera la moins grande possible. Pour qu'il en soit ainsi, le Gouvernement doit opposer rapidement une communication transparente, continue et proactive, en associant les professionnels de santé de proximité, mais aussi les jeunes générations. Cet effort de communication sur les effets secondaires et sur l'absence de collusion économique entre les laboratoires pharmaceutiques et le pouvoir, par exemple, permettra de convaincre. Il n'y aura pas de vaccination sans consentement ; c'est un prérequis non négociable : que les fervents opposants soient rassurés Nous regrettons cependant certaines postures politiciennes, qui, en mettant en scène sur la place publique des discussions au sein de la communauté scientifique, contribuent à l'affaiblissement de leurs institutions et donnent du crédit à ce phénomène de défiance. Le deuxième principe est la gratuité : le vaccin est un bien commun, garanti à tous. Aucun Français ne doit y renoncer pour des raisons financières ou territoriales. Ainsi, rappelons que le Gouvernement a budgété 1,5 milliard d'euros dans le PLFSS et que le Sénat a voté un amendement, porté par notre groupe, avec le soutien du Gouvernement, visant à fixer la TVA à 0 % sur les vaccins contre la covid-19. Oui, nous devons sécuriser la vaccination des plus précaires. malheureusement qu'ils seront difficiles à retrouver au moment de la seconde injection. Aussi, la mise en oeuvre d'une véritable initiative « d'aller vers » est indispensable. Le troisième principe, c'est la démocratie sanitaire. Les Français doivent être écoutés et associés à la stratégie vaccinale. À cet effet, deux instances ont été saisies

» et d'émettre des observations et des recommandations au Gouvernement. De plus, je remercie le Gouvernement d'avoir accepté que les parlementaires participent à cet effort de transparence, grâce à la création de la commission conduite par Cédric Villani. Le quatrième et dernier principe est la sécurité : la vaccination se fera dans le strict respect de toutes les règles qui encadrent l'utilisation des produits de santé dans notre pays. Si un vaccin est autorisé, c'est au terme d'une procédure rigoureuse et stricte d'essais aux échelles européenne et nationale. Mes chers collègues, l'objectif de la vaccination est clair : protéger les Français et protéger notre système de santé. Les résultats des études cliniques convergent pour démontrer que la vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et ses formes graves. Or réduire les formes graves, c'est diminuer non seulement la mortalité, mais également le risque de saturation de notre système de santé. Pour réussir, nous devons, avant toute chose, garantir aux Français le nombre de vaccins nécessaires le moment venu. Le 21 décembre, l'Agence européenne des médicaments se prononcera sur l'autorisation de mise en circulation sur le marché des vaccins. La décision d'autoriser un vaccin dépend bien d'une autorité indépendante européenne et d'autorités nationales, également indépendantes, comme la HAS, chargée de définir les publics prioritaires à vacciner. La responsabilité du Gouvernement est que tout vaccin mis sur le marché ait bien reçu toutes les autorisations nécessaires pour assurer une vaccination des Français en toute sécurité et garantir que lesdits vaccins soient acheminés rapidement. À ce jour, 200 millions de doses sont fléchées vers la France. Pour une campagne vaccinale optimisée, nous devons construire une logistique adaptée, afin de stocker et de déployer sur le territoire ces vaccins, qui présentent des caractéristiques particulières et différenciées. nous devons aussi vacciner en priorité les personnes pour lesquelles le virus est le plus dangereux, parmi lesquelles il ne faut pas oublier- vous l'avez dit, monsieur le ministre -les populations précaires, que l'on trouve souvent dans des milieux urbains considérés comme des déserts médicaux. C'est le rôle de la HAS que d'établir un ordre très précis des personnes à vacciner. Cette priorisation fait consensus et je ne pense pas qu'il faille revenir dessus. N'oublions pas que cette stratégie par phases et par ordre de priorité répond à une double volonté d'une part, réduire les hospitalisations et les décès ; d'autre part, maintenir les activités essentielles du pays, particulièrement celles du système de santé. Bien évidemment, la stratégie vaccinale vient compléter les dispositifs mis en place depuis le début de la pandémie. Parce que beaucoup ne sont pas considérés comme prioritaires et ne seront pas vaccinés avant des mois, les gestes barrières, le télétravail, le couvre-feu et toutes les mesures qui ont prouvé leur efficacité devront être maintenus ou adaptés dans le temps, avec beaucoup d'humilité, pour optimiser la protection de chacun. Une fois les vaccins mis sur le marché, nous entrerons dans la campagne de vaccination avec une seconde étape, celle de la vaccinovigilance, qui est indispensable pour suivre la distribution des doses vaccinales, afin que nous soyons capables d'en mobiliser de nouveau si besoin pour des personnes prioritaires. Il s'agit enfin de collecter des données en temps réel, et cela dès la première piqûre. C'est un arsenal complet qui va être déployé. Tous les échelons sont mobilisés pour garantir la plus grande transparence. Une cellule régionale de vaccination est mise en place au niveau de chaque Une collecte de donnée se fera à l'échelle régionale, avec les 31 centres régionaux de pharmacovigilance installés dans les hôpitaux. Ils recueilleront en temps réel les potentiels effets inattendus liés aux vaccins ou les cas dits « marquants », par exemple les problèmes cardiaques. produits de santé, l'ANSM, sera chargée, grâce aux remontées de terrain, de rendre public un rapport hebdomadaire sur les effets indésirables. Ces documents permettront de diffuser une information claire et accessible aux publics à toutes les phases de la campagne. Bien évidemment, tout cela ne se réalisera qu'avec la pleine mobilisation des professionnels de santé, des patients et des associations de patients. Nous aurons tous la possibilité de faire remonter ces informations grâce à un portail de signalement, qui, d'ici au lancement de la campagne, sera renforcé et promu auprès du grand public. Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des professionnels de santé. Pour autant, celle-ci ne sera possible que grâce à une nécessaire information du corps médical, claire et transparente, sur les types de vaccin, leurs modes de conservation et les populations destinataires. faudra surtout prévoir un statut juridique et assurantiel qui protège les médecins. Mes chers collègues, nous vivons une pandémie terrible, mais aussi une révolution scientifique extraordinaire. L'arrivée du vaccin marquera un tournant dans la lutte contre la covid-19. surmonter la défiance de tous, a dû s'administrer lui-même son propre vaccin. Aujourd'hui, en faisant confiance à la science et au monde médical, nous serons à la hauteur de la mission que notre mandat nous assigne,

Dans le contexte d'angoisse, de sacrifice et de colère de nos concitoyens provoqué par cette crise sanitaire et économique inédite, une stratégie vaccinale claire et précise est nécessaire pour redonner confiance à nos concitoyens. Alors que le Royaume-Uni a entamé, la semaine dernière, sa campagne de vaccination et que l'Allemagne a d'ores et déjà mis en place d'importants moyens logistiques, nous ne pouvions que nous interroger sur le retard de la France en la matière. Il a fallu attendre le 30 novembre pour que la Haute Autorité de santé publie ses recommandations et permette au Gouvernement d'en dégager une doctrine, alors que l'avis du conseil scientifique du 9 juillet pressait le Gouvernement d'agir dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, monsieur le ministre de la santé, il devenait urgent que la France se dote d'une stratégie de vaccination nationale qui permette d'établir clairement les conditions d'approvisionnement, de stockage, d'allocation, de distribution et d'administration du vaccin. Bien entendu, le déploiement de la vaccination doit viser en priorité les publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Le déploiement en trois phases proposé par le Gouvernement est judicieux pour permettre un accès équitable aux vaccins des personnes selon leur âge, leur comorbidité ou leur exposition. Néanmoins, le Gouvernement ne cesse de répéter qu'il a conduit une politique de préachat visant à sécuriser l'accès de la France aux vaccins en quantité suffisante. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite deux injections à quelques semaines d'intervalle. Pour autant, quelle sera la chronologie précise de ces livraisons ? De quelles garanties disposons-nous sur les commandes d'un point de vue logistique ? Nous pouvons nous inquiéter que, au pays de Pasteur, 61 % des citoyens aient annoncé, dans un récent sondage, n'avoir pas forcément l'intention de se faire vacciner. Ce chiffre édifiant repose en grande partie sur l'irresponsabilité dont quelques personnalités médiatiques ont fait montre en remettant en cause la crédibilité des discours scientifiques, ce qui alimente les fantasmes sur les futurs vaccins. Que n'a-t-on entendu de la part de spécialistes divers et variés, qui inondaient les informations de leurs avis dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas, comme la santé publique ? éminent réanimateur et dire des sottises sur l'attitude collective à adopter en réponse à une épidémie. Néanmoins, ces inquiétudes sont légitimes en l'absence d'une information complète sur les vaccins, au regard de la rapidité de leur développement, malgré les autorisations délivrées par les agences sanitaires européennes.

La question de la confiance est centrale ; elle doit être au coeur de cette stratégie. Les Français doivent comprendre que se faire vacciner est un acte citoyen pour parvenir de nouveau à vivre en société.

apparaît pertinent au regard de l'injonction de pédagogie et de clarté qu'exigent nos concitoyens. Il s'agit d'un acte fort en faveur de la démocratie sanitaire. Le professeur Alain Fischer a ainsi rappelé hier matin, lors de son audition par notre commission des affaires sociales, que les avis de ce conseil allaient être rendus publics. L'effort d'information et de transparence doit être ambitieux, pour inciter les Français à se faire vacciner. De même, je vous encourage à tabler au maximum sur une communication horizontale, plutôt que verticale, et à vous appuyer sur les relais importants que constituent les professionnels de santé et la société civile. Je tiens également à saluer le choix annoncé par le Gouvernement de laisser la vaccination facultative et gratuite, mais surtout de placer le médecin généraliste au centre de cette campagne. Les professionnels de santé seront en première ligne pour convaincre les patients du bienfait de cette vaccination. En effet, je le redis, seule la confiance pourra fonder le succès du déploiement de cette stratégie. Toutefois, les médecins restent surchargés. Aussi serait-il pertinent d'ouvrir le plus tôt possible aux pharmaciens et au personnel infirmier la possibilité de vacciner, comme c'est le cas pour la vaccination contre la grippe saisonnière, vaccination dont on peut se réjouir qu'elle ait nettement progressé cette année. ailleurs, il faut rappeler le succès de la coopération européenne en matière de stratégie vaccinale. La Commission européenne a ainsi engagé 2,7 milliards d'euros au sein de son instrument d'aide d'urgence pour financer les laboratoires les plus avancés dans leurs recherches. Cet investissement permet également de précommander des doses qui seront partagées entre les États membres selon des conditions tarifaires avantageuses. Enfin, nous avons affaire à une pandémie ; elle ne pourra donc être combattue qu'à l'échelle internationale. À cet égard, nous devons nous interroger sur la conception des vaccins comme biens communs universels, de manière à assurer un accès sûr, équitable et universel aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins en faveur des pays les plus pauvres. Nous devons en effet refuser toute compétition mondiale où la règle serait celle du chacun pour soi. L'initiative financière mondiale ACT a permis de mobiliser 2 milliards d'euros pour agir auprès des populations vulnérables et faciliter la recherche, ainsi que la diffusion du vaccin et des traitements. Ces discussions sur la solidarité internationale doivent être approfondies. Quels pays seront aidés et selon quelle chronologie ? Des doses leur seront-elles réservées ? ? Liberté de se faire vacciner ou non, égalité de l'accès au vaccin gratuit pour tous et fraternité envers celles et ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays développé et protecteur comme le nôtre : voilà les enjeux à considérer pour rester fiers de notre République. En résumé, monsieur le ministre, transparence et communication claire, sans bureaucratie excessive dans la transmission des décisions : voilà ce qu'il faut pour redonner confiance dans nos chercheurs, nos médecins

? J'étais ici le 9 novembre ! L'organisation de ce débat sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19 nous permet de prolonger les interrogations issues des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur la crise sanitaire. Alors que la pandémie de covid-19 a bouleversé la vie de toutes et de tous, l'arrivée de vaccins contre le virus est une excellente nouvelle. Cette nouvelle étape dans la lutte contre la covid-19 s'inscrit dans la stratégie définie, le 24 novembre dernier, par le Président de la République, Emmanuel Macron : « Tester, alerter, protéger, soigner. » Reste à conquérir l'adhésion de la population, sachant que seulement 41 % des Françaises et des Français auraient l'intention de se faire vacciner, selon un sondage Convaincus des bienfaits de la vaccination, nous partageons, monsieur le ministre, les recommandations de la HAS, qui n'est pas favorable à une vaccination obligatoire. Nous pensons en effet qu'il faut privilégier l'intelligence humaine sur les mesures coercitives qui seraient contre-productives. Il faut donc engager des moyens pour une véritable campagne de prévention sur la vaccination et associer les citoyennes et les citoyens aux décisions politiques. Les multiples scandales sanitaires- le Mediator, la Dépakine, le Distilbène, l'hormone de croissance, le sang contaminé et l'Isoméride, pour ne citer que quelques exemples -ont entraîné une méfiance d'une partie de la population envers les médicaments et les industriels. Comment peut-il en être autrement quand on voit les grandes puissances rafler plus de 6 milliards de doses de vaccins et n'en laisser que 500 millions pour le reste du monde ? Nous sommes non pas dans la coopération, mais dans la concurrence et le chacun pour soi Comment peut-il en être autrement quand les contrats commerciaux avec les Big Pharma sont totalement couverts par le secret des affaires ? Comment peut-il en être autrement quand règne une véritable opacité sur le prix auquel l'Union européenne achète ses stocks de vaccins ? La transparence doit s'imposer à tous les niveaux, y compris pour la composition des vaccins. La course contre le virus ne doit pas nous faire perdre de vue la sécurité sanitaire. Nous soutenons l'engagement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de publier, chaque semaine, un rapport sur les effets secondaires et indésirables signalés sur le vaccin. Afin de rassurer nos concitoyennes et nos concitoyens, nous vous suggérons, monsieur le ministre, de mettre en place un dispositif de vaccinovigilance consolidé. La stratégie vaccinale prévoit deux circuits de distribution : une centaine d'hôpitaux répartis dans chaque département et cinq plateformes nationales équipées de super-congélateurs. On nous dit que les généralistes auront un rôle pivot ; encore faudrait-il qu'ils possèdent les équipements nécessaires pour conserver les vaccins ! En effet, ni les hôpitaux, ni les Ehpad, ni les grossistes répartiteurs ne sont actuellement tous équipés de super-congélateurs, tant s'en faut. Selon notre groupe, l'achat de ces congélateurs doit se faire sur le budget de l'État et non sur celui de la Sécurité sociale ou des établissements eux-mêmes. Depuis l'annonce de l'arrivée des premières doses au début de 2021, une question se posait : quelles populations seraient prioritaires ? La HAS a tranché, en proposant cinq phases vaccinales, ce qui paraît adapté à la situation. Néanmoins, je souhaiterais vous faire part de plusieurs interrogations. Premièrement, dispose-t-on de suffisamment de personnel pour réaliser la vaccination ?

Quand on sait que le groupe pharmaceutique AstraZeneca a annoncé vendre son vaccin au prix coûtant de 4 euros, on peut s'interroger sur la portée des paroles d'Emmanuel Macron considérant que le vaccin contre la covid-19 est un bien commun de l'humanité, vendu à prix coûtant. À cet égard, je voudrais rappeler l'initiative citoyenne européenne portée par une large coalition de syndicats, d'ONG, de militantes et militants politiques, d'associations étudiantes et d'experts de la santé, qui vise à recueillir un million de signatures pour obtenir un accès équitable aux futurs vaccins et autres traitements pour pour toutes et tous en Europe et dans le monde, et pour lever l'opacité des négociations entre l'Union européenne et les laboratoires pharmaceutiques. On peut résumer cette campagne par la formule « ni profits ni monopoles sur la pandémie ». Je regrette vivement que le Sénat ait rejeté, la semaine dernière, notre proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux. C'était l'occasion de s'appuyer sur un outil public de production et de distribution des médicaments, ainsi que des vaccins à l'échelle nationale, mais

Je veux enfin attirer votre attention, monsieur le ministre, sur la stratégie de certains grands laboratoires, dont Sanofi : tout en recevant des fonds publics, ce laboratoire affaiblit au fil des ans ses activités de recherche et développement sur des thématiques essentielles,

En conclusion, si le vaccin n'est pas la solution miracle, c'est une pierre importante dans le combat que nous menons contre la pandémie. Aussi, ne manquons pas ce rendez-vous, mais tirons des leçons de ce que nous avons vécu avec les masques ou les tests

La question qui nous est posée est celle de la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19. La réponse est tout sauf simple, ce qui démontre l'importance des défis à relever. En effet, si nous construisons pas à pas des connaissances scientifiques, médicales et sociologiques, de simples îlots de certitudes au milieu d'un océan d'incertitudes et d'imprévus. D'une part, ce virus est nouveau ; bien que l'on connaisse mieux sa virulence et son pouvoir pathogène, il reste beaucoup à apprendre, notamment en clinique et en thérapeutique.

? Ce que nous savons, c'est combien cette maladie est grave, notamment pour les plus âgés et les plus fragiles. Nous savons aussi que les mesures barrières et le confinement sont efficaces. Nous savons enfin que, dès que l'on baisse la garde, l'épidémie reprend vite et fort ; l'actualité de ce jour le démontre Un vaccin efficace et aux effets secondaires limités est donc l'idéal attendu. Soyons réalistes : il va se passer encore un peu de temps avant que ce virus ne prenne la place qui doit être la sienne, celle d'un agent pathogène connu et contrôlé, avec lequel nous vivrons plus sereinement. Pour cela, le défi est d'agir individuellement et collectivement le plus efficacement possible, le temps que nous passions de l'inconnu à la connaissance. Dans cette stratégie, la vaccination est une clé essentielle. Pour autant, elle arrive dans un contexte d'incompréhensions et de doutes par rapport à la puissance publique et la science. La vaccination, qui est pourtant un formidable espoir, reçoit en effet un accueil mitigé de la part de nombre de nos concitoyens. ne pouvons, ni économiquement ni humainement, rater le rendez-vous de la vaccination, deux conditions s'imposent au Gouvernement pour que cette stratégie vaccinale soit une réussite dès sa première phase

C'est accepter de dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. C'est répondre à toutes les questions que nos concitoyens se posent de manière légitime. C'est aussi fournir, au fur et à mesure du déploiement de la vaccination, des points d'étapes de son avancement et de l'état des connaissances. C'est, enfin, éviter de tenir un discours pour ne pas avoir à tenir un autre. risques nouveaux, peut-être, parmi lesquels des effets secondaires rares qui ne pourraient se faire jour que quand un grand nombre de personnes seraient vaccinées. Il est donc essentiel que les données de la chaîne de pharmacovigilance et de la traçabilité des doses dispensées soient disponibles, actualisées, fiables et irréprochables. À ce titre, comme le préconise le rapport de l'Opecst, un site internet unique et ergonomique est vivement souhaitable. On pourrait y trouver l'avis des autorités sanitaires et scientifiques, nationales comme européennes, ou encore les études scientifiques au fur et à mesure de leur parution. Ce suivi est essentiel pour que chacun comprenne le processus et l'avancée de la stratégie jusqu'à la vaccination de la population générale, d'autant que nous aurons alors plusieurs vaccins différents. C'est à ce moment-là que l'adhésion des Françaises et des Français devra être la plus grande, dans l'espoir d'une immunité qui enraye la propagation du virus. La transparence, c'est aussi aborder la question de la nature et du montant des contrats conclus avec les laboratoires pharmaceutiques, en particulier la clause d'irresponsabilité, qui cristallise d'ores et déjà bien des suspicions. Outre cette transparence sur les contenus, un effort essentiel est à produire sur l'organisation des circuits de l'information. Depuis le début de cette crise, les querelles de plateaux alimentent les doutes ; la parole publique est elle-même source de confusion. La multiplicité des interlocuteurs produit des dissonances, parfois même des contradictions.

Il est temps de dire précisément qui fait quoi. Il est temps aussi de choisir qui informe, sur quoi, et comment. Bref, chacun son rôle : la parole publique doit être claire et lisible. Enfin, la transparence, c'est viser des publics et des canaux variés, c'est choisir prioritairement ceux qui, sur le terrain, seront les transmetteurs et les promoteurs privilégiés de la vaccination. Dans cette logique, le déficit d'information à l'égard des médecins est regrettable- on a pu le vérifier hier soir

car le colloque singulier entre le médecin et son patient sera un moment crucial dans l'adhésion à la vaccination. Les soignants dans les structures de santé et les pharmaciens sont eux aussi des rouages stratégiques d'information ; ils sont encore nombreux à devoir être convaincus. Il paraît d'ailleurs légitime de proposer dès à présent la vaccination à tous les soignants qui le souhaitent. Ce serait un acte positif d'exemplarité. Par ailleurs, nous ne saurions trop insister sur la nécessité de s'appuyer sur les associations de patients et d'usagers et de concevoir avec elles une stratégie de communication à destination des citoyens.

Ces questions de circuit et d'organisation de l'information doivent être réglées avant le début de la campagne vaccinale. Comme vous l'aurez compris, monsieur le ministre, cela doit passer, selon nous, par moins de verticalité et plus de proximité. Autrement dit, il s'agit de préférer la communication racinaire aux éclairs de Jupiter

Les vacciner, c'est les protéger. C'est aussi, en cas de recrudescence du virus, permettre aux hôpitaux d'accueillir tout le monde, en ayant protégé ceux qui étaient les plus vulnérables. Cette phase est donc un choix de raison, humainement et médicalement, mais il faudra très vite engager également la vaccination des personnes âgées à domicile.

autour des masques et des tests ont bien montré les limites de l'hypercentralisation. J'insiste vraiment, monsieur le ministre : tirez les enseignements des mois passés ! Nous attendons donc que cette organisation s'appuie sur les relais de terrain pour avoir la réactivité et l'agilité nécessaires. En amont, l'identification géographique des structures et du nombre de personnes à vacciner, en lien avec le nombre de doses disponibles, est une partie délicate de la chaîne. Intervient alors ce préalable essentiel qu'est le recueil du consentement éclairé des personnes. À ce sujet, l'orientation initiale était celle d'un consentement oral, auquel médecins et directeurs sont opposés : est-ce décidé ? Concernant les personnes âgées ne pouvant émettre un consentement éclairé, tuteurs, curateurs, tiers de confiance et familles doivent être identifiés dès à présent : ce sont eux qui prendront la décision de vaccination et devront être convaincus. Par ailleurs, les médecins lancent l'alerte sur leur responsabilité dans le cadre de cette campagne vaccinale : ils veulent se sentir juridiquement protégés, comme pour le H1N1. Un arrêté ministériel est ici nécessaire ; c'est vraiment un élément potentiellement bloquant ! Cruciale, parce que déterminante pour l'adhésion de la population générale, la réussite de cette première phase repose ainsi sur une logistique impeccable et complexe, que nous suivrons avec attention. le ministre, j'aimerais affirmer ici de manière claire et précise que nous accueillons avec espoir l'arrivée de la vaccination dans la stratégie globale de lutte contre la covid-19. Cet accueil s'accompagne d'une extrême attention et d'une particulière vigilance. Nous ne pouvons pas rater le rendez-vous de la vaccination : ce serait regrettable pour la lutte contre cette épidémie comme pour l'ensemble de la vaccination, avancée majeure dans la lutte contre un grand nombre de maladies.

Les vaccins sont une lueur dans une crise majeure. D'ici là, il faudra beaucoup d'écoute et de pédagogie pour maintenir la vigilance et l'adhésion aux mesures barrières et aux protocoles imposés, indispensables tant que le virus circule, ce

et le respect scrupuleux du rôle de chacun dans notre République. La parole

souhaitons de franchir cette épreuve sans dommage pour lui-même et ses proches. Faites-vous aussi notre messager, s'il vous plaît, auprès du préfet de police de Paris qu'il ait pour le chef de l'État l'indulgence qu'il n'a pas eue envers les Parisiens au printemps dernier, quand il a accusé ceux qui avaient été contaminés d'en être responsables en ayant enfreint les gestes barrières et le confinement, ce qui était très injuste.

plutôt me livrer à un exercice de mémoire. En effet, si le passé ne dicte pas l'avenir, du moins il l'éclaire. Rappelons-nous que notre pays, grâce à la vaccination, a éliminé des maladies

Notre époque n'accepte plus un tel rapport bénéfices-risques ; elle en demande un qui soit beaucoup plus net. C'est heureux, c'est le progrès, mais cela nous éclaire sur un point : ce n'est pas parce que de nouveaux outils comportent des risques qu'il faut les écarter.

La vaccination est donc un acte de santé publique qui permet aussi de lutter contre l'égoïsme et l'individualisme ; c'est un acte qui nous engage collectivement. Monsieur le ministre, vous pouvez être assuré de notre soutien dans la mise en oeuvre de cette stratégie de vaccination

à permettre au professeur Alain Fischer de mettre en application, à l'occasion de cette stratégie vaccinale, les dispositions qui étaient contenues dans le rapport de 2016. Il ne sert à rien de réinventer l'eau tiède tous les quatre matins ferions bien mieux d'appliquer les bonnes dispositions qui ont déjà été pensées et mûries. Je tiens à ajouter quelques mots,

et propositions que nous voulions partager avec vous, en attendant que le vaccin nous permette de mettre à l'abri les populations les plus vulnérables

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la stratégie vaccinale contre la covid-19 est un sujet qui soulève de nombreuses interrogations : comment, en effet, mettre en oeuvre cette vaccination au regard des règles actuelles et des besoins de la population ? La Haute Autorité de Santé a fondé ses recommandations sur une diminution de la morbi-mortalité liée à la covid-19, en se focalisant sur l'âge, puis sur la présence de facteurs de santé à risque. Dans la phase initiale, durant laquelle un nombre limité de doses sera disponible, deux populations apparaissent prioritaires, en raison de leur vulnérabilité et de leur exposition accrue au virus. Il s'agit des résidents d'établissements accueillant des personnes âgées et des personnels exerçant dans ces mêmes établissements. L'autorisation de mise sur le marché devrait être rendue par l'Agence européenne des médicaments le 21 décembre

Premièrement, qu'en est-il du consentement libre et éclairé des personnes qui se feront vacciner ? Je rappelle que les conditions du consentement sont prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information étant délivrée au cours d'un entretien individuel. Le consentement libre et éclairé à la vaccination contre le covid-19 suppose donc que les patients soient informés au préalable, par leur médecin traitant, de l'efficience du vaccin, de ses éventuels effets indésirables et des contre-indications.

Avez-vous prévu que la phase de recueil du consentement et la vaccination se fassent de façon distincte, conformément à ce que prévoit l'article 1111-2 du code de la santé publique ? Le cas échéant, un début de vaccination contre le covid-19 dès la fin du mois sera-t-il compatible avec la législation actuelle ? en ce qui concerne la première phase de vaccination dans les Ehpad, 30 % des établissements ne disposent pas de médecin coordinateur et, dans beaucoup d'autres, le médecin ne passe dans l'établissement qu'une fois par semaine, ce qui risque de compliquer l'organisation de la vaccination.

Plusieurs raisons plaident en faveur d'une vaccination s'appuyant sur les médecins généralistes, qui ont la confiance de leurs patients, ainsi que sur les infirmiers libéraux et les pharmaciens. Comment envisagez-vous de construire l'organisation de la vaccination de masse ? Y aura-t-il des régions ou des départements prioritaires ? Quel sera le rôle des préfets et des élus locaux ? Quelle est la composition du comité d'élus locaux que vous envisagez de réunir tous les quinze jours, et quel sera son rôle ? Enfin, j'appelle l'attention du Gouvernement sur la situation des 3,8 millions de Français qui vivent dans des territoires sous-dotés en médecins généralistes, soit 6 % de la population. Il ne serait pas acceptable que les Français habitant dans les déserts médicaux pâtissent, durant cette campagne de vaccination, du faible nombre de professionnels de santé.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis de longs mois, l'épidémie de covid-19 mobilise sans discontinuer nos professionnels de santé, met à terre notre économie et démoralise notre nation. La perspective d'un vaccin est donc un fantastique espoir, qui semblait hors de portée il y a quelques mois encore. La recherche a été rapide et constitue un élément de satisfaction, dans une période qui en compte peu. À l'heure où cet espoir se fait jour et où d'autres pays s'emploient déjà à le matérialiser, j'observe que le débat se focalise sur la supposée réticence des Français à se faire vacciner. Prenons garde que, à faire tourner en boucle cette défiance, elle ne finisse par s'auto-entretenir. La couverture vaccinale des Français n'est pas très bonne, il est vrai, mais celle des enfants l'est, et le passage à onze vaccinations obligatoires n'a pas soulevé la levée de boucliers annoncée. Pour réussir la stratégie vaccinale, il faut relever de nombreux défis, qui sont avant tout logistiques : la mise à disposition de vaccins en nombre suffisant- c'est là la vraie question conservés dans de bonnes conditions et administrés aux bonnes personnes et par les personnels les plus appropriés. Souvenons-nous de l'échec de la campagne de vaccination contre la grippe A. Notre collègue Alain Milon, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale de l'époque, déplorait « l'incompréhension face à une campagne de santé publique à laquelle n'étaient pas associés les médecins ». Il pointait là une condition majeure du succès d'une stratégie vaccinale : le médecin traitant est central pour la prise en charge de ses patients. Les généralistes, les pédiatres, les sages-femmes, les infirmiers et, d'une façon générale, l'ensemble du premier recours,

Prenons l'exemple du comité scientifique sur les vaccins covid-19, créé au premier semestre 2020 : il ne comportait alors aucun médecin généraliste et, de façon tout aussi surprenante, il ne comprenait aucun représentant des usagers du système de santé

fondée sur un rationnel scientifique puissant. La HAS a déjà produit deux avis sur une stratégie vaccinale contre le covid-19, en juillet et en octobre 2020 ; notre commission a entendu sa présidente hier.

dont on saisit mal l'articulation avec les agences sanitaires et les instances déjà mises en place, même si je tiens à saluer la clarté de l'intervention du professeur Fischer, hier, devant la commission des affaires sociales. Devant cette profusion d'avis, quelle instance scientifique allez-vous finalement écouter pour arrêter votre stratégie ? Je terminerai par la sécurité : c'est en rassurant nos concitoyens sur cet enjeu que nous gagnerons leur confiance. Leurs interrogations sont légitimes face à des techniques vaccinales nouvelles. À cet égard, notre système de pharmacovigilance, pour assurer une veille permanente des moindres incidents, sera déterminant. Quels moyens comptez-vous y Plutôt que de laisser les théories complotistes les plus fantaisistes empoisonner le débat public, nous devons les combattre avec détermination, science à l'appui. Dans cet exercice, notre meilleur allié, une fois encore, est toute la communauté de professionnels en santé, qui a la confiance des Français. C'est en garantissant leur adhésion à la stratégie que nous pourrons les convaincre. J'ai bien compris l'étalement en différentes phases, qui semble lié, pour partie, à l'impossibilité de garantir des vaccins en nombre suffisant. Mais alors que beaucoup de Français sont impatients,

J'attends de ce débat que vous nous montriez comment vous entendez en tenir compte. La parole

Structure commune au Sénat et à l'Assemblée nationale, sous la double présidence de Gérard Longuet et de Cédric Villani, l'Opecst « a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique, afin d'éclairer ses décisions.

dont j'avais eu l'honneur d'être la rapporteure avec deux collègues députés, Cédric Villani et Jean-François Eliaou. Pour alimenter le débat d'aujourd'hui, l'Opecst a désigné quatre rapporteurs : deux sénatrices- Sonia de La Provôté

Premièrement, ce vaccin constitue une avancée scientifique majeure. Le SARS-CoV-2 provoque des réactions très hétérogènes selon les personnes. Nous savons aussi qu'il tue, l'âge étant le principal facteur de risque. Dans l'urgence, le vaccin protège les plus fragiles et évite la survenue de la maladie. Nous pensons que le vaccin Pfizer-BioNTech, qui sera le premier disponible, présente une balance bénéfices-risques favorable, pour protéger notamment les personnes âgées en leur évitant de développer une forme grave de la maladie.

En résumé, si l'intérêt individuel du vaccin est d'ores et déjà certain, l'intérêt collectif, quant à lui, l'est moins. Deuxièmement, afin d'assurer le succès de cette protection vaccinale,

Nos recommandations sont simples, et il est impératif que la première phase de la vaccination soit réussie pour favoriser l'adhésion de la population, ce qui suppose de ne pas se précipiter. Nous pensons aussi que les professionnels de santé qui le souhaitent et les personnes au contact de publics fragiles devront pouvoir être vaccinés rapidement, si ce n'est prioritairement. Il conviendra surtout de s'appuyer, en confiance, sur les professionnels de santé de ville, en les informant largement de tous les aspects de la stratégie de vaccination et en prenant rapidement l'arrêté qui permettra l'intervention de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'Oniam, afin que Il faudra aussi que le traçage des vaccinations opérées soit efficace, ne serait-ce que pour réaliser la seconde injection, indispensable pour assurer l'efficacité du premier vaccin, Le carnet de vaccination électronique est un outil intéressant, qui pourrait être mis en oeuvre dans la stratégie vaccinale. Troisièmement, la rapidité avec laquelle les sociétés américaines ont pu mettre au point un vaccin innovant doit nous interroger sur notre capacité à soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine médical. S'il est tout à fait positif que les pays européens aient choisi de négocier collectivement l'achat de vaccins avec les grands laboratoires, il est aussi manifeste que nous ne disposons pas des outils permettant d'investir massivement dans le développement des médicaments stratégiques ou innovants. La, ou Barda, américaine, qui a investi 10 milliards de dollars, sous la forme de partenariats public-privé, pour la mise au point de vaccins, permet aujourd'hui aux États-Unis de bénéficier de livraisons prioritaires et de conditions de prix plus favorables. L'Europe devra s'en inspirer. Quatrièmement, et surtout, il nous faut gagner la confiance de nos concitoyens. Cette confiance est possible : quelque 15 millions de vaccins contre la grippe ont été administrés dans notre pays en un temps record, à savoir moins de six semaines ! Il faudra répondre aux craintes qui s'expriment dans ce contexte de crise avec un nouveau virus, en explicitant l'analyse bénéfices-risques dans la concertation, la publication des travaux devant aussi contribuer au climat de confiance. Cette dernière ne sera possible que grâce à une totale transparence

des personnes ou les aider dans les transports. Le choix des cibles vaccinales suscite un véritable débat, que vous ne trancherez pas en tant que sénateurs et que je ne trancherai pas comme ministre. C'est la Haute Autorité de santé, qui

pas. Je dirai simplement que je ne porte pas un regard critique sur ceux de nos concitoyens qui ne se sentent pas à ce stade à l'aise concernant le vaccin. D'ailleurs, le Président de la République a annoncé lui-même que la vaccination ne serait pas obligatoire. Il ne s'agit pas de forcer les gens à accepter le vaccin le vaccin ou de considérer que ceux qui ont peur, qui s'inquiètent ou qui s'interrogent auraient tort de le faire. Nous sommes un peuple doté d'un esprit critique, et c'est aussi ce qui fait de nous un grand peuple scientifique. Saint Thomas disait : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». probable que le niveau de confiance augmentera dans la population à mesure que la campagne de vaccination progressera, mais je ne reproche jamais à quelqu'un d'avoir peur d'un traitement que l'on veut lui prescrire.